Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. Monsieur le Premier ministre,

Il est accompagné par nos collègues Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées,

Dans un contexte international d’une exceptionnelle gravité, et face aux incertitudes pesant sur l’avenir du lien transatlantique, un forum tel que l’Assemblée parlementaire de l’Otan, qui offre aux parlementaires des 32 pays de l’Alliance un

À ce titre, l’Assemblée parlementaire de l’Otan, dont nous célébrons cette année le soixante dixième anniversaire, représente un outil précieux et efficace de la diplomatie parlementaire et met en exergue

chers collègues, en votre nom à tous, permettez moi de souhaiter à M. Perestrello la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française.

qui remplace M. Philippe Bas, nommé au Conseil constitutionnel. Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Nous aurons l’occasion d’échanger entre Normands,

souveraineté industrielle et numérique, les États Unis reviennent sur la suspension de leur aide à l’Ukraine. Un espoir fragile de cessez le feu avec la Russie se profile, mais rien n’est encore gagné. On ignore ce que seront les contreparties auxquelles l’Ukraine devra consentir. On ignore pour l’heure ce que sera la position de la Russie. Cette séquence diplomatique, dont nous espérons qu’elle sera un premier pas vers une résolution du conflit, ne doit pas nous détourner de nos responsabilités. Pouvoir compter sur notre propre défense n’est pas une option, mais une nécessité. Notre groupe sait clairement ce qu’il veut : une Europe forte, capable de défendre ses intérêts stratégiques propres. Une telle ambition européenne sera servie d’abord par une ambition nationale française et par un effort d’investissement d’ampleur. Nos entreprises de défense s’organisent ; c’est vrai, notamment, dans le département dont Monsieur le ministre, si vous souhaitez que les Français consentent un tel effort d’investissement, une transparence totale s’impose. À l’évidence, si l’on ne veut pas augmenter la pression sur nos finances publiques, nos possibilités sont limitées. Mobiliser l’épargne des Français peut s’entendre, à condition que cela soit consenti. Allez vous créer un livret dédié au financement de notre défense ? Quand comptez vous faire des annonces concrètes à cet égard ? Laisser les Français dans l’incertitude, c’est faire le lit des opposants à cet objectif vital.

Monsieur le sénateur Daubet, la question est sérieuse, et nous y travaillons très activement depuis que le Président de la République, dans son discours de la Sorbonne, a souhaité que l’Union européenne acquière son autonomie stratégique. Un réveil est en train de se produire à la suite des événements tragiques qui se déroulent en Ukraine et qui nous obligent dorénavant à prendre en main notre destin, y compris en matière de défense. Nous y travaillons à tous les niveaux.

afin que les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permettra d’assurer la sécurité de notre pays et de l’ensemble de l’Union européenne. La parole

Monsieur le ministre, après la tentative de racket sur les terres rares, l’humiliation du président Zelensky dans le Bureau ovale, la trahison de l’arrêt de l’aide militaire, l’Ukraine vit un nouveau revirement américain avec le rétablissement de l’aide et la proposition d’une trêve. Soit. C’est une bonne nouvelle, mais comment l’Ukraine peut elle avoir confiance dans l’administration Trump, dont la conception du droit consiste à ce que les règles ne s’appliquent que lorsqu’elles servent ses intérêts ? Face à ces pressions et à cette instabilité, l’Ukraine a plus que jamais besoin du soutien politique, économique et militaire de l’Europe. Certes, nous avons pris des mesures fortes : une aide financière supérieure à celle des États Unis et l’utilisation des intérêts des avoirs russes gelés. Mais aujourd’hui, face à l’urgence et à l’incertitude, se pose la question de l’utilisation des 210 milliards d’euros d’avoirs gelés en Europe pour financer l’effort de défense ukrainien, pour prix de la résistance et d’une paix juste. sein du Gouvernement, émettent des réserves juridiques ou économiques sur cette saisie, quand d’autres s’appuient sur le droit coutumier international pour la justifier. Au delà du débat juridique, quel est le plus grand risque ? L’utilisation de ces avoirs ou la déstabilisation de l’ensemble du continent européen ? Est ce à l’agresseur ou aux citoyens européens de payer ? Ma question est simple : le Gouvernement compte t il porter cette exigence de justice devant le prochain Conseil européen ?

Monsieur le ministre, les Ukrainiens attendent des gestes forts de la part de l’Europe et la Russie ne peut se prévaloir d’une règle de protection légale de ses actifs alors que M. Poutine piétine le droit international. L’utilisation de ces fonds contribuerait à inverser le sentiment d’impunité de la Russie, et pourrait même être un élément de négociation. Permettez moi de citer le Président de la République : « L’Europe doit retrouver le goût du risque, de l’ambition et de la puissance. » Passons des paroles aux actes

mon groupe a toujours condamné, sans hésitation, l’agression odieuse de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, la violation du droit international perpétrée par la Russie et les crimes de guerre commis par son armée. Nous appelons à une paix juste, garantissant la sécurité du pays agressé et écartant toute capitulation. Depuis lundi, sous la pression d’un Trump pressé de mettre fin à ce conflit pour faire des affaires librement, des négociations ont commencé. Nous regrettons, comme beaucoup, que l’Europe subisse le tempo du président américain et n’ait pas été à l’initiative. Nous sommes à un tournant, face à cet axe qui se met en place entre Trump et Poutine. Comment y répondre ? En accumulant les armes toujours plus, encore et encore ? En suivant Mme von der Leyen, qui affirme que « le temps est venu d’assurer la paix par la force » ? Qui peut croire que les peuples ont à gagner dans cette course folle aux armements ? Pouvez vous nous indiquer, monsieur le ministre, en quoi le plan d’économie de guerre de 800 milliards d’euros présenté par Mme von der Leyen représente un gage de paix pour l’avenir ? Le Président de la République indiquait, surjouant les menaces et les peurs : « Il faudra des réformes, des choix, du courage.

L’effort de guerre, madame la sénatrice, est surtout un effort pour la paix. Dans un monde devenu plus dangereux, nous sommes convaincus que l’Europe doit se protéger. Cette protection doit être autonome, indépendante des États Unis, et nécessitera de mobiliser des moyens nouveaux.

Ensuite, vous dénoncez la trahison de Trump. Mais, demain comme aujourd’hui, c’est l’Otan sous commandement américain que vous financerez et surarmerez toujours plus. S’émanciper de Trump et des USA, c’est sortir, dans un premier temps, du commandement intégré de l’Otan !

Notre pays a aujourd’hui pris conscience de la menace que fait peser le narcotrafic sur sa sécurité intérieure. L’administration pénitentiaire a un rôle fondamental à jouer dans le combat engagé par l’État contre ce phénomène. L’objectif est clair : empêcher les détenus, qu’ils soient prévenus ou condamnés, de poursuivre leurs activités criminelles depuis leur cellule. La désignation des deux premiers établissements pénitentiaires de haute sécurité marque votre volonté d’agir, monsieur le ministre d’État, et d’agir vite. Le choix de Condé sur Sarthe, dans l’Orne, après celui de Vendin le Vieil, dans le Pas de Calais, traduit une véritable reconnaissance du professionnalisme de ses agents pour la prise en charge des détenus les plus dangereux. le cas pour Vendin le Vieil, votre décision nécessitera des moyens complémentaires, au sein de l’établissement comme à l’extérieur. Au sein de l’établissement, la nécessité de renforcer les effectifs est une évidence. Surveillants sur la coursive, équipe locale de sécurité pénitentiaire ou encore renseignement il nous faut trouver les moyens pour attirer des profils expérimentés, sans évidemment déshabiller le centre de détention d’Argentan, situé à quarante kilomètres, et déjà en manque de personnel. À l’extérieur de l’établissement, quel sera l’impact du choix de Condé sur Sarthe sur l’activité du tribunal judiciaire d’Alençon et, surtout, sur les forces de sécurité intérieure ? La question du prêt de main forte par la police ou la gendarmerie pour les extractions que nous n’aurons pas réussi à éviter, celle de la protection des agents pénitentiaires et de leurs familles contre les risques de pression, ou encore celle de la lutte contre les activités illicites qui auraient été attirées par la présence à Condé sur Sarthe de ces détenus hors norme, ne sauraient être traitées à moyens constants, c’est à dire avec ceux qui sont présents dans un département rural comme l’Orne. Aussi, monsieur le ministre, pouvez vous rassurer les Ornais sur le nécessaire renforcement des moyens de l’État pour assurer la réussite du projet de prison « anti narcos » à Condé sur Sarthe, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement ? La parole

J’ai malheureusement constaté que le groupe socialiste et le groupe écologiste n’avaient pas voté favorablement en commission des lois… J’espère qu’ils le feront la semaine prochaine, pour le bien de l’administration pénitentiaire. bien de l’administration pénitentiaire. Je suis heureux de saluer la présence dans nos tribunes des auditrices et des auditeurs de la huitième promotion de l’Institut du Sénat. Sur l’initiative de notre ancien collègue Jean Léonce Dupont, le bureau du Sénat avait décidé en 2015 de mettre en œuvre ce programme de formation, en vue de mieux faire connaître les modalités de fonctionnement et les enjeux de notre démocratie parlementaire à des personnalités d’horizons géographiques et professionnels très divers.

Monsieur le ministre, notre devoir, depuis le 24 février 2022, est de rendre certain l’échec de l’agression russe en Ukraine. Et depuis que les Américains ont élu un impérialiste autoritaire totalement erratique, aux mains d’un autocrate impérialiste froidement calculateur, notre devoir est d’être en mesure, en tant qu’Européens, d’assurer notre sécurité et de défendre nos valeurs de manière autonome aujourd’hui et demain. Or, depuis la semaine dernière, on entend que les nécessaires investissements dans la défense se feront sans taxer les riches, c’est à dire sur le dos du climat, des services publics, du vélo et même des retraites. C’est terriblement dangereux et complètement idiot

directement l’agression poutinienne contre nous ! La réalité, c’est que la transition énergétique n’est pas en concurrence avec la défense : elle fait partie intégrante de notre arsenal pour battre Poutine. C’est la même chose pour la justice sociale. Quand la classe moyenne

que de laisser Poutine gagner

sous nos yeux, l’ordonnancement du monde est bouleversé et notre sécurité remise en question. Dans ce contexte inédit depuis plusieurs décennies, il nous faut plus que jamais nous adapter et prendre des décisions à la fois fermes et fortes. Le Président de la République et le Gouvernement ont fixé un objectif nouveau, auquel je souscris, de hausse de notre effort militaire au delà de la trajectoire de la loi de programmation militaire. Cet effort pèsera sur le budget de l’État pour l’achat des matériels et des équipements militaires. Il nécessitera un financement privé spécifique de nos entreprises pour leur permettre d’adapter leurs capacités de production. Cet effort se ferait sans augmentation d’impôts, sans toucher à nos dépenses sociales et – vous venez de le dire – sans augmenter notre dette. augmenter notre dette. Pouvez vous nous dire quelles seront les sources et les modalités de financement de cet effort de défense tout à fait inédit ? À quelle hauteur nouvelle

Madame la ministre, c’est la deuxième fois que j’interviens sur le dossier de l’enseignement primaire à Wallis et Futuna. Je remercie l’État d’avoir enfin pris l’engagement, cinquante cinq ans plus tard, d’intégrer le personnel enseignant et non enseignant dans la fonction publique d’État.

tout en garantissant le respect de nos spécificités locales. Le rapport de l’inspection générale de l’administration a été rendu. Sous le pilotage du préfet et de la vice rectrice, les groupes de travail ont réuni tous les acteurs locaux : les élus, les représentants des chefferies coutumières, la mission catholique, les syndicats et les parents d’élèves. Ainsi, le consensus recherché par le Gouvernement a été trouvé. je vous remercie d’avoir été particulièrement attentive à ce dossier, ce qui a permis la tenue de la réunion interministérielle définitive le vendredi 7 mars

et pour garantir la mise en place concrète du statut de l’enseignement primaire à Wallis et Futuna, avant l’été 2025 ? La parole

je vous remercie de votre question et d’avoir souligné que nous avons pris ce dossier à bras le corps depuis mon arrivée au ministère. Oui, l’État va tenir sa parole en ce qui concerne le statut des enseignants du premier degré à Wallis et Futuna. Le protocole signé en juillet 2023 est à cet égard fondamental. L’évolution du statut des enseignants doit permettre d’assurer l’égalité territoriale et également être un levier pour la réussite des élèves. Tout comme en métropole ! J’y suis attachée, comme l’ensemble des acteurs du territoire. À la suite de ce protocole, vous l’avez rappelé, une mission interministérielle a rendu ses conclusions, qui prévoient des mesures tant législatives que réglementaires. J’ai l’ambition que ce travail se concrétise rapidement. Il a donc été fait le choix d’un projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnance,

Comme l’État s’était engagé à être prêt pour la rentrée du 17 février dernier, une mesure compensatoire sera mise en place pour la période allant de cette date à l’entrée en vigueur effective de la réforme, afin qu’aucun enseignant ne soit lésé par ce décalage.

La réforme sera bientôt entre les mains du Parlement. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation lors de son prochain examen au Sénat. La parole est à M. Marc Laménie, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Pour l’organisation des jeux Olympiques, la reconstruction de Notre Dame et maintenant celle de Mayotte, à chaque fois, le Gouvernement a fait voter au Parlement un texte d’exception. En France, en 2025, dès que l’État veut entreprendre un projet, il est obligé de s’autoriser lui même par la loi à déroger aux lourdeurs administratives qu’il impose aux citoyens et aux acteurs économiques que sont les entreprises, les agriculteurs et les indépendants. Une autre solution serait d’alléger cette lourdeur administrative pour tout le monde, en réduisant radicalement ces normes, puisque l’État peut s’en passer. Le président Olivier Rietmann, sénateur de Haute Saône, nous alertait déjà sur

et plus que le budget du ministère de la défense. Un premier projet de loi de simplification de la vie économique a été présenté par un gouvernement précédent au mois d’avril 2024. La Haute Assemblée l’a examiné en responsabilité, et il sera prochainement examiné par l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, ma question est simple : quel est le programme de travail

et nos concitoyens de vivre correctement leurs rapports avec nos administrations. En tant que ministre chargé de la simplification, je ferai dans les semaines à venir un certain nombre de propositions qui viendront s’ajouter au projet

voir ce que l’administration peut faire à la place de nos concitoyens dans le cadre des démarches administratives qu’ils réalisent. Ensuite, je compte sur l’ensemble des bonnes volontés au Parlement

L’Alaouite au tombeau, le Chrétien à Beyrouth. » Malheureusement, l’Histoire bégaie encore une fois, que ce soit pour les Chrétiens et Yézidis massacrés en Irak et en Syrie par Daesh, les Kurdes par la Turquie, les Juifs par le Hamas, les Arméniens d’Artsakh par l’Azerbaïdjan, les Européens par le totalitarisme islamique et les vagues d’attentats, et désormais, encore, les minorités en Syrie. En effet, le massacre, ces derniers jours, de milliers de civils, d’hommes, de femmes, chrétiens et alaouites, par des islamistes de toutes origines, nous le démontre de nouveau. Pourtant, lorsque ces derniers prirent le pouvoir en décembre dernier, leur chef Jolani prétendait que tous les Syriens étaient frères. Dès lors, la communauté internationale réunie sous l’égide du président Macron se précipitait pour soutenir la transition politique en Syrie. En effet, Jolani, pour reprendre la formule de Gilles Kepel, « djihadiste relooké par les turco qatari », n’était plus considéré comme un sanguinaire, mais comme un combattant de la liberté, puisqu’il portait une cravate et une barbe bien taillée. Pourtant, ce loup islamiste déguisé en agneau démocrate a refusé de serrer la main d’une femme, la ministre allemande en visite en Syrie avec notre ministre M. Barrot. C’est vrai ! Dès 2014, j’avais déjà alerté, aux côtés de François Fillon, sur la disparition de ces populations autochtones devenues minoritaires, victimes de ces crimes contre l’humanité et de génocide, notamment depuis 1915. Comme en Irak ou en Artsakh, la France assiste encore impuissante à une épuration ethnique, revendiquée par les Frères musulmans. Ne laissons pas la France faillir à son devoir historique et moral de protection des minorités ! Aussi, monsieur le ministre, alors que l’Union européenne s’est précipitée pour rencontrer Jolani, que compte faire la France pour que les pays européens parlent d’une même voix et agissent enfin pour protéger ces minorités persécutées en voie d’extinction ?

des exactions perpétrées ces derniers jours en Syrie. Il s’agit de crimes inacceptables que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Tous leurs auteurs devront être jugés Il n’y aura pas de justice sans que toute la lumière soit faite sur les événements tragiques qui ont eu lieu. Nous n’avons jamais eu ni naïveté ni complaisance à l’égard du nouveau pouvoir syrien. Nous avons exprimé auprès du ministre des affaires étrangères des autorités intérimaires syriennes, M. Chibani, notre indignation collective et l’exigence de protéger toutes les populations, à quelque communauté Nous condamnons également les tentatives de déstabilisation de la Syrie par des groupes proches du régime d’Assad, peut être appuyés par des ingérences étrangères qui ont lancé ce bain de sang. Nous prenons note Nous prenons note de l’annonce par les autorités intérimaires syriennes de la mise en place d’une commission d’enquête et d’un comité de la préservation de la paix civile. Alaouites, Chrétiens, Kurdes, Druzes, Sunnites, toutes les composantes du pluralisme syrien doivent trouver leur place et être traitées à égalité dans la nouvelle Syrie. L’accord politique conclu lundi entre les nouvelles autorités syriennes et nos partenaires kurdes des Forces démocratiques syriennes est un signe positif. La lutte contre le terrorisme islamiste et l’extrémisme doit aussi se poursuivre. À Paris, le 13 février dernier, la communauté internationale a exprimé conjointement ces principes et ces attentes, qui ont été entendues et endossées par les autorités syriennes. Il s’agit maintenant, si l’on veut éviter que la Syrie ne retombe dans l’horreur et la guerre civile de les mettre en œuvre sans délai. Il faut conclure ! La France ne ménagera aucun effort dans cette perspective. Valérie Boyer, pour la réplique. Monsieur le ministre, comment faire confiance à Jolani ? Comment éviter la solution finale, l’extermination totale de ces minorités

pour que la langue du Christ soit encore parlée par les Araméens, qui sont en voie d’extermination. Il faut conclure ! Monsieur le ministre, il ne faut pas les abandonner.

300 d’entre eux ont entamé une grève de la faim pour alerter sur la précarité dans laquelle ils sont placés. En effet, alors que, selon les mots du Président de la République lui même, « ils tiennent […] à bout de bras nos services de soins

Pour certains s’ajoute une précarité administrative, puisqu’ils sont astreints à renouveler chaque année, voire tous les six ou trois mois, leur autorisation de séjour. Enfin, pour obtenir l’autorisation de plein exercice et être inscrits au tableau de l’ordre des médecins, les Padhue doivent valider des épreuves de vérification des connaissances (EVC) particulièrement sélectives, puis effectuer un parcours de consolidation de deux ans. Les résultats de la session 2024 des EVC, parus le 31 janvier dernier, ont suscité une forte colère. Seulement un peu plus de 3 000 postes ont été pourvus, alors que 4 000 étaient ouverts par décret. Alors que les fédérations de Padhue dénoncent des critères d’admission opaques et arbitraires,

vous avez noté leur importance pour notre système de soins, ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent. Quand allez vous enfin proposer des mesures concrètes

jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre système de santé. Nombreux dans les hôpitaux publics, ils pallient souvent le manque de médecins, notamment dans les spécialités et les territoires en tension. Pourtant, leur situation administrative reste précaire, marquée par des procédures de régularisation longues et complexes ainsi que par une reconnaissance professionnelle inégale sur tout le territoire national. Depuis la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances, ils dénoncent par la voix de leurs syndicats une sélection qu’ils jugent inéquitable et incohérente. D’une part, le nombre de postes finalement pourvus est inférieur à celui qui était initialement ouvert. Certaines filières, pourtant en tension, sont particulièrement touchées : en médecine générale par exemple, 563 candidats ont été admis sur 826 postes ouverts ; et alors que la santé mentale est une priorité nationale, seuls 39 praticiens ont été admis sur 263 postes. D’autre part, les critères d’admissibilité semblent avoir varié selon les spécialités au gré des jurys. Certains candidats n’ont pas été admis avec une note supérieure à 10, tandis que d’autres, avec une note inférieure, l’ont été dans des filières différentes. Cette situation singulière est d’autant plus incompréhensible que ces médecins exercent dans nos hôpitaux depuis des années dans des conditions salariales souvent précaires, alors même qu’ils pallient la pénurie médicale qui frappe notre pays. Le Président de la République s’était engagé à régulariser ces professionnels en exercice. Pourtant, aujourd’hui, ces praticiens se sentent abandonnés face à cette situation qui compromet non seulement leur avenir professionnel et celui de leurs familles, mais aussi la qualité et la continuité des soins prodigués aux patients. Monsieur le ministre, que comptez vous faire pour répondre à la colère et au sentiment d’injustice exprimés par ces praticiens essentiels au fonctionnement de notre système de santé ?

Je vous remercie,

comment la France, qui a joué un rôle important dans la reprise du processus de reconstruction, compte t elle s’impliquer ? Peut on faire confiance au président par intérim sans jouer les idiots utiles de l’un ou de l’autre des prédateurs régionaux ?

je l’ai dit, la France condamne toutes les exactions contre les civils, quelles que soient les communautés visées et quels que soient leurs auteurs, groupes affiliés au régime de Bachar el Assad ou groupes terroristes. Il s’agit de justice, mais aussi de l’avenir de la Syrie. Nous n’avons eu de cesse de le répéter, ce pays ne pourra retrouver sa stabilité et sa prospérité sans un processus politique qui garantisse la sécurité et les droits de toutes les communautés. Je pense en particulier à la sécurité contre le terrorisme ou à la prolifération des armes chimiques. La lutte contre le terrorisme passe d’abord par le respect des droits et des intérêts des Kurdes en Syrie et par la destruction des stocks d’armes chimiques du régime. Les résultats obtenus lundi avec les Kurdes de Syrie sont très encourageants, et ont été suivis par un accord hier avec les Druzes. Par ailleurs, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques va pouvoir se déployer en Syrie pour détruire les stocks du régime de Bachar el Assad, qui constituent une menace pour la sécurité internationale. Ce travail doit se poursuivre parce qu’en Syrie se joue une partie de notre sécurité. Il va de soi que nous ne pourrons pas accepter de nouvelles levées de sanctions si nous n’avons pas de garantie que les exactions ne resteront pas impunies. Enfin, la France suit avec préoccupation les développements dans le Golan. Nous appelons donc Israël à la retenue. Toute action militaire unilatérale en Syrie ferait le jeu d’acteurs à l’agenda déstabilisateur, au premier rang desquels l’État islamique. La parole

Madame la ministre de l’agriculture, le 20 février dernier, la direction générale de la concurrence de la Commission européenne a sollicité la direction générale de l’alimentation de votre ministère pour qu’elle réponde à un questionnaire sur les financements publics des laboratoires départementaux d’analyses.

le rappelle, le groupe Eurofins, porteur de la plainte Aprolab, est une entreprise du CAC 40, installée au Luxembourg, dont les dirigeants habitent en Belgique et qui a défrayé la chronique dans plusieurs dossiers récents ; cela pourrait justifier de s’intéresser de plus près à ses pratiques. Madame la ministre, vous savez l’importance du rôle des laboratoires départementaux d’analyses dans le maillage sanitaire français et leur implication essentielle dans la gestion des crises récentes, comme celles du covid 19, de la grippe aviaire, de la fièvre catarrhale ovine ou encore de la maladie hémorragique et épizootique des bovins. Dans ces conditions, quelles actions quelles actions comptez vous engager pour permettre à nos laboratoires publics d’analyses, qui ont démontré leur efficacité et leur réactivité, de continuer d’exercer sereinement leurs missions au service de notre agriculture, de notre environnement, de notre santé et de notre souveraineté alimentaire ?

année durant laquelle l’association des laboratoires privés Aprolab a déposé une plainte auprès de la Commission européenne. Cette plainte ciblait, vous l’avez dit, les compensations attribuées aux laboratoires départementaux d’analyses par les conseils départementaux et qui, selon le plaignant, faussaient le coût des analyses dans le domaine concurrentiel privé. Cette procédure a été suspendue en 2020 par la Commission européenne elle même, à la faveur de la recherche d’une solution amiable entre les autorités françaises et les laboratoires du groupement Aprolab. Cette solution consistait à mettre en place des mandats de services d’intérêt économique général, chantier conduit à son terme quatre ans plus tard, avec l’appui politique du Gouvernement. Néanmoins, malgré les engagements pris, le plaignant estime dorénavant que des laboratoires visés dans la nouvelle plainte continuent de percevoir des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, en particulier de la part des conseils départementaux, sous forme de subventions d’équilibre. La Commission européenne a donc interrogé la France le 20 février dernier à propos de ces nouvelles plaintes. Mes services Mes services techniques et juridiques travaillent activement, en collaboration avec les laboratoires concernés et les représentants des collectivités territoriales, pour répondre à la Commission européenne.

relatif à la baisse brutale et rétroactive des soutiens aux petites et moyennes installations solaires en toiture continue de provoquer colère et incompréhension.

De même, les particuliers qui se sont tournés vers l’autoconsommation, une démarche vertueuse qu’il convient d’encourager, risquent de ne pouvoir faire ces investissements coûteux en effet, dans le secteur de l’autoconsommation, le taux réduit de TVA de 5,5 % n’entrerait en vigueur qu’en octobre prochain, alors même que les aides gouvernementales ont pris fin le 1 février dernier ! N’est ce pas incohérent ? ailleurs, voilà moins d’un an, était signé avec l’État un Pacte solaire destiné à soutenir le déploiement et l’industrialisation photovoltaïque en France. Ce pacte est il passé aux oubliettes ?

J’en veux pour preuve l’approche de la lutte contre les stéréotypes de genre, omniprésente dès la maternelle, qui prend systématiquement la forme d’une contestation des représentations du féminin et du masculin. En outre, le projet introduit, dès la classe de cinquième, la dissociation artificielle entre sexe et genre. Nous ne croyons pas qu’il appartienne à l’école de la République de créer un doute identitaire chez nos adolescents sur des réalités biologiques établies, alors même que cette période de la vie est marquée par une construction de soi qui qui doit être sécurisée par des repères clairs et bienveillants. À l’inverse, plusieurs enjeux fondamentaux de la vie affective et relationnelle sont complètement occultés de ce nouveau programme. L’enseignement de l’éducation à la sexualité impose de transmettre des informations objectives et adaptées à l’âge des élèves, dans le respect du principe de neutralité. Vous avez annoncé deux jours de formation au profit des intervenants du programme destiné aux jeunes de 3 à 18 ans, sur un sujet éminemment sensible et intime. C’est irréaliste ! Qui assurera ces séances ? Comptez vous faire appel au planning familial ? Que dire enfin de l’exclusion incompréhensible et inacceptable des parents de l’information préalable sur les séances d’Evars, alors que ces derniers doivent être pleinement informés et associés au contenu des interventions ? Nous ne pouvons accepter que l’éducation sexuelle soit le cheval de Troie de la théorie du genre et du « transactivisme » à l’œuvre dans nos écoles. Face à ces dérives, nous exigeons que soient enfin garantis un respect strict du principe de neutralité, un renforcement de la prévention contre les dangers réels et le rétablissement du droit à l’information des parents.

et à la sexualité. Nous, non ! Ce sont évidemment des sujets sensibles, qui doivent être abordés avec beaucoup de rigueur et de discernement. C’est précisément la raison pour laquelle, en juin 2023, alors que j’étais Première ministre, j’avais demandé au ministre de l’éducation nationale de saisir le Conseil supérieur des programmes,

Les experts du Conseil supérieur des programmes ont ainsi veillé à la progressivité et à l’adéquation du programme, en fonction de l’âge et de la maturité des élèves.

soyons clairs, les familles seront bien associées, informées du contenu de ces programmes comme de tous les autres, notamment lors des réunions parents professeurs de début d’année. la sénatrice, selon moi, garantir à chaque enfant une éducation au respect, au consentement, à l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est lui donner les clés pour se protéger et grandir en confiance ;… Il faut conclure ! … cela relève de notre responsabilité collective et c’est ce à quoi s’emploie ce programme d’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité.

pour la première fois en France, une étude a porté sur l’incidence des cancers chez les adolescents et les jeunes adultes de 15 à 39 ans, dans dix neuf départements. Les résultats de ces travaux, connus depuis le 3 mars dernier, ont révélé une hausse constante de l’incidence de plusieurs types de cancers entre 2000 et 2020. Sur cette période, les glioblastomes ont augmenté de 122 %, les carcinomes du rein de près de 90 % et les liposarcomes de 74 %. Bien que n’évoluant pas à la même vitesse, la tendance observée pour les carcinomes colorectaux, les cancers du sein et les lymphomes de Hodgkin n’en demeure pas moins préoccupante. J’ajoute, comme le démontrent plusieurs études récentes, que la progression de certains cancers précoces n’est pas propre à notre pays. Selon un article paru dans le en 2023, le nombre de nouveaux cas chez les moins de 50 ans est passé de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019. Face à cette situation alarmante, il semble indispensable de mieux comprendre les facteurs de risque et les dangers liés à certaines expositions, et d’y sensibiliser les jeunes adultes.

prévoyez vous d’affiner les stratégies de prévention et de faciliter l’accès précoce au dépistage,

dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal, je souhaitais m’abstenir. Par ailleurs, lors du scrutin public n° 222 sur l’article 1de la même proposition de loi, Mme Corinne Bourcier souhaitait s’abstenir.

L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales. Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.

La parole est à M. le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.

chose promise, chose due ! Voilà six semaines, je m’engageais à ce que le Gouvernement prolonge le dispositif des concours Talents jusqu’en 2028. Aujourd’hui, nous allons, je l’espère, graver cet engagement dans le marbre de la loi.

La prorogation des concours Talents est d’abord motivée par la situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il est nécessaire d’adopter ce texte au plus vite, à la fois pour sécuriser juridiquement les places des concours existants

exige pour faire vite de faire conforme. À cet égard, je remercie les sénateurs de la commission des lois, qui, sensibles à nos arguments et à l’impérieuse nécessité d’aller vite, ont adopté le texte sans modification et à l’unanimité la semaine dernière. Nos débats d’aujourd’hui ne sont pas uniquement d’ordre juridique, car cette proposition de loi témoigne, en réalité, d’un enjeu bien plus important : la manière dont un État fort recrute ses meilleurs agents publics. Avec ce texte, nous abordons deux concepts qui me semblent essentiels pour l’avenir de la fonction publique, à savoir l’attractivité et la méritocratie républicaine. À sa manière, cette proposition de loi consacre, au fond, le droit de chacun peu importe d’où il vient – d’aspirer aux plus grandes responsabilités administratives dans notre pays. Pour attirer les talents, il faut aller les chercher partout où ils sont, dans tous nos territoires, en métropole comme dans nos outre mer. En somme, il faut savoir recruter des talents issus de tous milieux sociaux. C’est dans cette optique que le dispositif des prépas Talents a été mis en place et que le Gouvernement a créé des concours externes, les concours Talents, permettant à l’État de former les cadres de demain. Signe d’ouverture, de démocratisation et de succès du dispositif, les toutes dernières places offertes à ces concours l’ont d’ailleurs été dans les outre mer, territoires auxquels je sais

De la montée en puissance de nos capacités de défense au renforcement d’une stratégie nationale de résilience en passant par la mise en œuvre du plan d’adaptation du territoire au changement climatique – Christophe Béchu a porté ce sujet lorsqu’il était ministre –, nous aurons de plus en plus besoin besoin d’ingénieurs supplémentaires, à la tête bien faite, dans les rangs de la fonction publique. Enfin, la prolongation de l’expérimentation des parcours et des concours Talents, ainsi que leur sécurisation juridique jusqu’en août 2028, permettra à l’ensemble des parlementaires et au Gouvernement de disposer de données consolidées sur plusieurs années et d’un bilan pour acter ou non, avec recul, l’intérêt de pérenniser ce dispositif qu’il nous faut encore mieux faire connaître au grand public. À cet égard, je recevrai dans les prochaines semaines l’association La Cordée afin que nous puissions valoriser le dispositif et les parcours des élèves au sein du service public.

permanent et de concertation. Nous le devons aussi à nos institutions. Nous aurons donc l’occasion – j’en suis sûr – de travailler ensemble sur de nombreux textes d’initiative parlementaire, que je soutiendrai, pour améliorer la fonction publique dans son ensemble et le quotidien de celles et de ceux qui veulent servir la France. La parole

unanimement favorable, je relève que le parcours législatif de ce texte aura été particulièrement rapide. Déposé le 19 décembre dernier par la députée Florence Herouin Léautey, il a été voté par l’Assemblée nationale le 18 février commission des lois l’a adopté, sans modification, mercredi dernier, selon la procédure de législation en commission. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 20 janvier. De façon logique, cette accélération du calendrier est liée à la nécessité de proroger dès que possible l’expérimentation des concours du plan Talents du service public, alors que celle ci a pris fin brutalement le 31 décembre dernier. Bien sûr, l’urgence à légiférer face à laquelle nous sommes aujourd’hui placés résulte directement du manque d’anticipation dont a fait preuve le pouvoir exécutif : celui ci a laissé l’expérimentation aller à son terme sans remettre au Parlement le rapport d’évaluation qui avait été prévu dans la loi pour le 30 juin 2024 au plus tard. Certes, le gouvernement actuel n’est pas responsable des soubresauts politiques des mois derniers, mais il n’en est pas moins regrettable de devoir se prononcer dans l’urgence sur la prorogation de cette expérimentation. Il est à espérer que cette situation ne se reproduira pas et qu’il sera donné au Parlement la possibilité de décider en amont et en connaissance de cause de la pérennisation ou non de ce dispositif. Ces remarques de méthode étant faites, j’en viens au contenu de la proposition de loi adoptée par la commission des lois. Comme vous le savez, l’expérimentation des classes préparatoires et des concours Talents a débuté en 2021, à la suite de l’ordonnance du 3 mars 2021, qui découlait elle même de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi, les classes prépas Talents ont succédé aux classes préparatoires intégrées. Accessibles sur dossier et après un entretien de motivation, elles visent à permettre à des étudiants issus de classes socioéconomiques défavorisées de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour préparer les concours de la fonction publique, en particulier les six concours externes spéciaux dits Talents. ont été mis en place pour l’accès à cinq écoles de service public formant des cadres d’emploi de catégorie A+ dans les trois versants de la fonction publique : l’Institut national du service public, pour l’accès à la voie générale, l’Institut national des études territoriales, pour la formation d’administrateur territorial, l’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour la formation de directeur d’hôpital et de directeur d’établissement sanitaire, social et médico social, l’École nationale supérieure de la police, pour la formation de commissaire de la police nationale, et l’École nationale d’administration pénitentiaire (Enap), pour la formation de directeur des services pénitentiaires. Le nombre de places offertes par année aux lauréats des concours Talents est compris entre 10 % et 15 % du nombre de places ouvertes au titre du concours externe classique d’accès à l’école concernée. Aussi bien le jury que les programmes et les épreuves sont identiques à ceux du concours externe Dans la mesure où l’expérimentation s’est éteinte du jour au lendemain, sans qu’une pérennisation du dispositif ait été proposée, une forte insécurité juridique pèse sur les concours Talents de la session 2025, comme M. le ministre l’a rappelé. Les écoles de service public ont d’ailleurs abordé l’organisation de cette session de manière variable : l’ENSP et l’INSP ont pris un arrêté d’ouverture de concours à l’été 2024, l’Inet et l’EHESP au début de l’année 2025. l’Enap, elle a fait le choix de ne pas ouvrir de concours Talents au titre de cette session. Les calendriers des épreuves sont eux mêmes variables : les épreuves d’admissibilité du concours de commissaire de police nationale ont eu lieu dès le mois de janvier celles du concours de l’INSP auront lieu dans deux semaines et les premières épreuves de l’Inet, de l’EHESP et de l’ENSP sont, quant à elles, prévues au mois de juin De plus, un contentieux est en cours devant le Conseil d’État dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté d’ouverture du concours Talents pour l’accès à l’INSP. Comme vous l’aurez compris, mes chers collègues, il est indispensable de sécuriser les concours Talents de la session en cours. cours. Au delà, il paraît également opportun de proroger pour trois années supplémentaires cette expérimentation, soit jusqu’en août 2028 comme le prévoit le texte, de manière à disposer de suffisamment de recul et de données en vue de réaliser un bilan étayé.

De surcroît, cette évaluation est d’autant plus indispensable que le périmètre de l’expérimentation aura lui même été élargi à de nouvelles écoles, comme le prévoit l’article 1 du texte. Celui ci ouvre en effet la possibilité de créer une voie Talents dans les écoles formant les militaires, en particulier pour l’accès au corps des ingénieurs de l’armement. la commission partage l’objectif de favoriser une plus grande diversité sociale et territoriale au sein de la haute fonction publique, y compris dans les grands corps techniques, elle a souligné les spécificités inhérentes aux règles de recrutement des membres de ces corps, qui limitent fortement la portée d’éventuels concours Talents. La commission a toutefois adopté cette disposition, dont le bilan devra être soigneusement établi le moment venu. Au regard de l’urgence à redonner aux concours Talents une base légale, la commission des lois a adopté sans modification cette proposition de loi, que je vous invite à voter ainsi. Au delà de ce texte, j’invite le Gouvernement à mener une réflexion de fond sur la nécessité de renforcer l’attractivité de la fonction publique auprès de l’ensemble des jeunes et d’agir en faveur de l’égalité des chances le plus en amont possible. La parole est à Mme Patricia

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd’hui à nous prononcer sur la prorogation de l’expérimentation des concours Talents pour l’accès à certaines grandes écoles de service public. Il s’agit d’un dispositif essentiel, qui vise à renforcer l’égalité des chances et à lutter contre les déterminismes sociaux en ouvrant davantage la haute fonction publique à la diversité des parcours et des origines. Depuis leur mise en place en 2021, ces concours s’adressent aux étudiants boursiers issus des classes préparatoires Talents, lesquelles offrent un accompagnement renforcé aux jeunes aux ressources limitées. L’objectif est clair : permettre à chacun, quelle que soit de suivre sa vocation et d’accéder aux plus hautes responsabilités publiques. Ce n’est pas une remise en cause du principe du mérite, bien au contraire ! Il s’agit de s’assurer que les talents de notre pays s’expriment pleinement, sans être bridés par des inégalités de départ. Pourtant, au 31 décembre dernier, ce dispositif est arrivé à échéance sans que le rapport d’évaluation prévu ait été rendu dans les délais. Cette situation a entraîné une insécurité juridique pour les concours Talents de la session 2025, qui avaient déjà débuté dans certains établissements. Une intervention législative urgente s’est donc imposée afin d’éviter que les candidats ne se retrouvent privés d’une opportunité pour laquelle ils se sont investis pleinement. C’est tout l’objet de cette proposition de loi, adoptée sans modification en commission. Elle prévoit la prorogation du dispositif jusqu’au 31 août 2028, afin que nous puissions disposer d’un bilan complet et fiable sur les effets réels le report de la remise du rapport d’évaluation au 31 mars 2028, ce qui permettra d’analyser la réussite et l’intégration des lauréats dans la fonction publique ; la sécurisation des concours Talents ouverts dès 2025 afin de lever tout risque juridique pesant sur les épreuves en cours ; l’extension de l’expérimentation à certains corps d’ingénieurs de l’État, dans le but d’élargir encore le champ des des opportunités offertes. Ce texte répond donc à une double nécessité : garantir la continuité du dispositif et une évaluation approfondie avant toute décision de pérennisation. La commission des lois du Sénat a ainsi validé sans modification la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, car elle est consciente de l’importance de donner aux jeunes concernés une visibilité et une sécurité indispensables pour leur avenir. Comme nous le savons, les grandes écoles de service public sont marquées par une homogénéité Si nous voulons une haute fonction publique qui reflète la diversité et les réalités de notre société, alors nous devons continuer à ouvrir des voies d’accès qui garantissent à tous les talents, sans distinction d’origine, la possibilité de s’engager au service de l’intérêt général. Le groupe RDPI soutiendra donc cette proposition de loi avec conviction, car elle traduit des engagements républicains forts : l’égalité des chances et la promotion d’une fonction publique plus inclusive, plus ouverte et plus représentative de notre pays. La parole

depuis maintenant plusieurs décennies, notamment grâce aux travaux menés en matière de sociologie, il n’est plus possible d’ignorer les lacunes structurelles en matière d’accès à l’enseignement et leurs conséquences à long terme. La notion de « capital culturel » a largement mis en lumière le déterminisme auquel pouvait se heurter un enfant ou un jeune adulte de cet héritage transmis par le milieu social et familial valent tout particulièrement pour les études supérieures. Aussi la seule proclamation du principe d’égalité ne suffit elle Cette prise de conscience de l’inégalité des chances en matière d’éducation doit inciter les pouvoirs publics à œuvrer à un décloisonnement. Si l’égalité des chances est essentielle partout, elle l’est d’autant plus pour accéder à notre fonction publique : une administration ne saurait être le reflet imparfait de la société qu’elle sert. Toute forme d’isolement risquerait de lui faire perdre ce qui fait sa légitimité : sa capacité à comprendre, à représenter et à protéger chacun de nos concitoyens. C’est à cette ambition qu’a répondu la mise en place des concours Talents du service public en 2021. Par cette innovation bienvenue, nous avons su reconnaître que l’excellence ne naît pas toujours dans les mêmes cercles, que le potentiel n’a pas d’adresse et que, souvent, il suffit d’un coup de pouce et d’un cadre adapté pour qu’une vocation fasse son œuvre. En offrant un accompagnement renforcé, ces classes préparatoires ont ouvert les portes des grandes écoles de la fonction publique à des étudiants issus de milieux défavorisés, prouvant que la réussite est une question non pas d’origine, mais d’opportunité. pourtant que cette belle dynamique a été brutalement stoppée. La fin de cette expérimentation, programmée au 31 décembre 2024, a laissé derrière elle un vide juridique et une incertitude pesante. Que deviennent les candidats qui ont travaillé sans relâche pour préparer ces concours ? Quelle réponse leur donner alors que certaines écoles ont déjà commencé les épreuves tandis que d’autres hésitent, paralysées par l’absence de cadre légal ? Laisser les choses en l’état reviendrait à trahir la promesse faite à ces jeunes, en refermant les portes que nous venons de leur ouvrir. Dans ces circonstances, la proposition de loi que nous examinons n’est pas qu’un simple ajustement technique, elle est une nécessité. D’abord, elle permet de prolonger l’expérimentation jusqu’en 2028, évitant ainsi l’interruption brutale d’un dispositif qui commence à peine à porter ses fruits. l’adoption de cette proposition de loi sécurisera les concours déjà ouverts, la fin de l’expérimentation ayant plongé la session 2025 dans l’incertitude. En assurant la continuité du dispositif, ce texte vise à protéger les candidats d’une annulation injuste et à garantir l’équité des épreuves. Tout à fait. Nous comprenons évidemment les difficultés institutionnelles qui ont fait obstacle à une prolongation du dispositif par le Gouvernement durant l’hiver dernier. pouvons malgré tout regretter que le rapport qui devait être remis à l’été 2024 n’ait jamais été publié. Enfin, en étendant l’expérimentation à d’autres corps de la fonction publique, cette proposition de loi élargit encore le champ des possibles pour ceux qui, jusque là, en paraissaient exclus. En somme, cette proposition de loi ne corrige pas seulement une faille juridique, elle conforte un outil essentiel pour rendre la fonction publique plus accessible et plus représentative de la diversité de notre société. Toutefois, ce texte ne résout pas tout. Une sensibilisation dès le secondaire permettrait de montrer à tous ces jeunes qui n’osent même pas rêver de la fonction publique que, avec du travail, ces métiers sont aussi les leurs. les publics ciblés sont souvent mal informés de l’existence des prépas Talents, ce qui limite leur portée. Assurer la promotion de ces dispositifs est l’unique moyen de donner aux futurs candidats l’envie de se projeter L’égalité des chances n’est pas seulement un concept abstrait. Elle est une idée qui, lorsqu’elle prend forme, change des destins, transforme des vies et enrichit notre République.

le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à diversifier le recrutement dans la haute fonction publique. Fort du constat hélas ! peu encourageant

Au cœur de cette réforme, le dispositif des filières Talents avait pour objet de faciliter l’accès des étudiants issus de milieux modestes, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, à cinq grandes écoles de service public, en leur réservant 10 % à 15 % des places offertes aux concours externes.

placé les candidats ayant déjà commencé la préparation des concours de l’année 2025 dans une situation d’incertitude quant au maintien de ces derniers. Fort heureusement, la mobilisation politique et transpartisane sur ce sujet ainsi que la volonté du Gouvernement, représenté par M. le ministre Laurent Marcangeli, que je tiens à saluer amicalement,

La prépa Talents n’est pas seulement un programme d’accompagnement, c’est un véritable levier de transformation sociale répondant au droit de chaque élève talentueux d’intégrer la fonction publique, de servir l’État et de contribuer à la richesse et à la diversité de nos institutions.

Bien qu’il ne puisse à lui seul remédier au défaut d’égalité des chances dans la fonction publique, ce dispositif diversifie sans conteste les origines géographiques des lauréats, répondant ainsi aux enjeux d’attractivité et de méritocratie qui doivent prévaloir.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

nous, voire impensable, de nous opposer à l’objectif d’égalité des chances dans l’accès aux grandes écoles de la fonction publique. Cependant, il ne faudrait pas que cette prorogation nous dispense d’une réflexion plus large et plus approfondie sur l’efficacité réelle du dispositif.

Nous sommes confrontés à un vide juridique alors même que des étudiants se sont préparés pendant des mois, voire pendant des années, pour ces concours. En tout état de cause, il nous paraît incohérent de passer d’un vide juridique à une prorogation automatique, sans réelle analyse de fond.

à celui de passer un concours. Elle se joue bien plus tôt, dès le collège et le lycée, notamment dans l’orientation scolaire et les choix d’études. Si nous nous contentons de mesures tardives, comme celles qui sont proposées le dispositif des prépas de ne toucher qu’une petite partie de la population estudiantine. L’égalité des chances, c’est d’abord offrir à tous les élèves, indépendamment de leur origine sociale ou géographique, des parcours d’éducation qui leur permettent d’accéder aux filières qui sont ici visées. L’accès aux grandes écoles et à la fonction publique est la résultante d’un parcours qui doit commencer bien avant Nous devons donc repenser l’éducation en amont, dès les premières étapes du parcours scolaire, en facilitant l’accès à des formations préparatoires adaptées, à des soutiens spécifiques et à une meilleure orientation dès le plus jeune âge. Faut il se satisfaire d’un dispositif qui ne concerne de fait qu’un nombre restreint d’étudiants ? Ne devrions nous pas réfléchir à des mesures plus ambitieuses, intervenant bien plus tôt, j’y insiste, dans les trajectoires scolaires ? Ce n’est qu’au travers d’un changement global, de l’école primaire au lycée, que nous pourrons véritablement offrir à chacun les mêmes chances de réussir ces concours. Un autre point mérite notre attention : l’extension du dispositif aux corps techniques d’encadrement supérieur de l’État. Si l’intention est louable, la réalité est plus nuancée. Les voies de recrutement dans ces corps sont très spécifiques, et l’ajout d’un concours Talents risque de n’être qu’une mesure symbolique sans effet réel sur la diversité des recrutements.

George Orwell montre comment le soulèvement démocratique des animaux au sein d’une ferme bascule progressivement vers un régime autoritaire. Les cochons, doués d’une intelligence supérieure, forment rapidement une élite et asservissent les autres animaux et les droits universels originellement proclamés sont bientôt réduits au seul commandement suivant : « Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d’autres. La situation de l’élite administrative française est à l’image de cette parabole. En théorie, le recrutement par concours place tous les candidats en situation d’égalité. Mais, en pratique, les différences de capital social entre les candidats favorisent certains les Parisiens représentent 2,5 % des étudiants, mais un tiers des admis dans les grandes écoles ; quant aux enfants des classes supérieures, singulièrement ceux des hauts fonctionnaires, ils y sont eux aussi surreprésentés. Les mécanismes de reproduction sociale par le biais du concours sont bien connus.

C’est le fameux arrêt. Or personne n’ignore ici l’influence des anciens élèves de l’ENA dans la conduite des affaires du pays. Ce phénomène va croissant avec le prestige entourant l’école : il est plus marqué encore pour l’INSP, la nouvelle école d’administration, que pour l’école nationale supérieure de la police. Certaines études récentes montrent que les chances d’intégrer l’ENA sont multipliées par 330 si le père du candidat en est lui même un ancien élève. telle situation n’est pas digne d’une grande démocratie. Il nous appartient donc de veiller à réduire les barrières administratives et sociales qui bloquent l’accès aux carrières publiques les plus prestigieuses. C’est pourquoi nous voterons cette proposition de loi qui vise à pérenniser l’expérimentation des classes préparatoires Talents mise en place en 2021. La proposition de loi de la députée Florence Herouin Léautey pallie ainsi les manquements du Gouvernement, qui n’a pas honoré son obligation d’informer le Parlement sur le bilan de l’expérimentation. Elle protège en outre les élèves admis dans les classes préparatoires spécifiques. Nous la soutenons donc sans réserve. Il importe toutefois de rappeler que ce dispositif ne permettra pas à lui seul de restaurer l’égalité des chances entre candidats en matière de carrières publiques. L’intégration dans ces grandes écoles clôt en réalité des parcours universitaires exemplaires, à l’université et surtout dans d’autres écoles déjà sélectives : l’ENS (École normale

Seules des réformes structurelles, comme l’instauration d’une allocation universelle d’études destinée à l’ensemble des étudiants, sur le modèle de ce qui existe dans les pays scandinaves et de l’allocation déjà versée aux étudiants normaliens, pourraient aboutir à une réelle égalité des chances.

Il y développe l’idée que la surproduction d’élites dirigeantes serait la cause de crises, voire de l’effondrement des sociétés, et ce en raison de la compétition qu’une telle surproduction ferait naître entre les cadres dirigeants. Dans le même temps, une récente étude de France Stratégie montre que 15 % des postes ouverts aux concours de la fonction publique n’ont pas été pourvus en 2022.

Nous restons fidèles à une vision claire, celle d’un service public de qualité, au service de tous, doté des moyens de fonctionner. La parole

alors que les enfants d’ouvriers représentaient 19,6 % de la population active française en 2019, ils ne constituent que 5 % des promotions des écoles de la haute fonction publique pour les années 2020 et 2021. Ce n’est en définitive guère mieux qu’il y a trente ans, lorsque, fille d’un ouvrier et d’une employée et première bachelière de la famille, j’entrais à Science Po Paris. Ces chiffres édifiants montrent combien, dans notre République, une forme de reproduction sociale continue de limiter les chances de nombreux jeunes, en particulier de celles et ceux qui sont issus des milieux les plus modestes. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutient de longue date toutes les initiatives favorisant non seulement l’égalité des chances, mais l’égalité réelle. La démocratisation des parcours éducatifs – de tous les parcours – ne s’oppose pas, selon nous, à l’excellence. Au contraire, elle la bonifie, parce que la diversité – sociale, géographique, académique – des profils dirigeants est créatrice de valeur, dans le secteur privé

Ces dispositifs sont des leviers indispensables pour permettre à des étudiants d’accéder à des métiers et à des écoles dont leurs parents comme eux mêmes ignoraient sans aucun doute l’existence jusqu’alors, la même occasion, de se mettre au service de l’intérêt général. C’est dans le cadre du plan Talents du service public et par l’ordonnance du 3 mars 2021 que les concours Talents ont été institués de manière expérimentale, pour trois ans, de relever la proportion d’élèves issus des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées dans les cinq écoles qui mènent aux trois versants de la haute fonction publique, l’INSP, l’Inet, l’EHESP, l’ENSP et l’ENA.

Malgré cela, aucune initiative gouvernementale nouvelle n’a vu le jour : ni évaluation en bonne et due forme et dans les délais utiles ni prolongation ou pérennisation de l’expérimentation.

Et c’est finalement l’initiative parlementaire qui a pris le relais, grâce à Florence Herouin Léautey et aux députés socialistes. Leur proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale le 19 décembre 2024 et que nous examinons aujourd’hui, a donc pour objet de revenir en trois points sur l’ordonnance de 2021 : prorogation de l’expérimentation des concours Talents,

Au regard de l’urgence qu’il y a à consolider la base légale des concours pour la session 2025, au regard aussi de l’attente angoissée des étudiants et de leurs familles, le groupe socialiste se joint en séance, comme il l’a fait en commission, au souhait d’un vote conforme, donc d’une entrée en vigueur au plus vite de la nouvelle ordonnance. Bien sûr, la prolongation des prépas et concours Talents ne suffira pas à elle seule à renverser des mécanismes de reproduction sociale encore profondément ancrés dans notre système éducatif et professionnel. Cette proposition de loi constitue néanmoins un pas utile vers un modèle plus inclusif, afin que chaque jeune, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, bénéficie de véritables chances d’accès aux fonctions d’excellence, y compris publiques.

l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose : « Tous les citoyens étant égaux [aux] yeux [de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Le législateur savait écrire… Exactement ! La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de concrétiser ce principe méritocratique auquel nous sommes tous attachés. Mais, pour obtenir une véritable égalité des chances, il ne suffit pas de dire à nos jeunes : « Les portes de nos écoles sont ouvertes ! » Il faut faire davantage pour ceux d’entre eux qui, justement, sont les plus défavorisés leur donner un coup de pouce. Tel est l’objet de ce texte. Je me réjouis qu’il soit examiné dans un esprit consensuel, bien au delà des clivages partisans : venant du Sénat, cela n’a rien d’étonnant.

Initialement conçu pour ne plus être applicable après le 31 décembre 2024, le programme Talents est donc prorogé jusqu’au 31 août 2028. En conséquence, la proposition de loi reporte au 31 mars 2028 la remise au Parlement par le Gouvernement du rapport d’évaluation de l’expérimentation. En deuxième lieu, il élargit la voie des concours Talents aux concours permettant l’accès aux écoles assurant la formation de militaires, afin d’y inclure l’accès au corps des ingénieurs de l’armement, ce qui est fondamental dans le contexte actuel.

traduit notre engagement à tous en faveur de l’égalité des chances, qui donne à chacun la possibilité de réussir en fonction de son mérite. Il faut rappeler cette vérité souvent oubliée l’État a besoin de tous les jeunes talentueux, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, et la fonction publique doit refléter la diversité de notre pays. mon propos sans saluer la qualité du travail de notre rapporteure, notre collègue Catherine Di Folco. Cette proposition de loi va en réalité bien au delà de la seule prolongation d’un dispositif elle relève un véritable défi, celui du renforcement de la méritocratie républicaine par l’édification d’une fonction publique plus représentative de l’ensemble de notre société.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité

madame la présidente,

transposent strictement le champ d’application de la directive NIS 2, en précisant les seuils à partir desquels les entreprises sont considérées comme des entités essentielles ou importantes. La rédaction se fonde, conformément à l’article 2 de la directive, sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne qui définit les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Comme la directive vise les grandes et moyennes entreprises, la rédaction actuelle du

pour l’article 8 qui définit les entités essentielles, le périmètre est celui des grandes entreprises, c’est à dire les entités qui ne relèvent pas de la catégorie des moyennes entreprises au sens de la définition de l’Union. La rédaction est donc proposée les entités essentielles sont les entreprises qui appartiennent à des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros et dont le bilan annuel excède 43 millions d’euros.

à la menace cyber. Par ailleurs, les communautés d’agglomération ont, en moyenne, une plus grande maturité en matière de numérique et de sécurité des systèmes d’information. Ainsi, 60 % des 229 communautés d’agglomération ont bénéficié d’un parcours de cybersécurité de l’Anssi et ont par conséquent d’ores et déjà accompli des progrès importants de sécurisation de leurs systèmes d’information. Elles auront donc des efforts moindres à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par la loi. Limiter le statut d’entité essentielle à certaines communautés d’agglomération serait risqué au regard du niveau de protection et du principe d’égalité. plusieurs communautés d’agglomération au profil démographique très proche, voire similaire, seraient alors soumises à des niveaux d’exigences différents. À titre d’exemple, la communauté d’agglomération du Grand Sénonais rassemble 60 000 habitants.

Il nous semble plus sécurisant pour les EPCI concernés, notamment pour la planification des investissements en matière de cybersécurité, d’être fixés dès l’adoption de la loi sur leur éventuel assujettissement, plutôt que de voir celui ci modifié en fonction de la population de la commune centre. L’objectif de massification de la cyberdéfense porté par la directive peut passer, pour les collectivités territoriales, par un effort et une incitation à la mutualisation de leurs systèmes d’information afin qu’elles puissent plus facilement répondre aux exigences.

ne comprenant pas au moins une commune dont la population est supérieure à 30 000 habitants. Il s’agit, dans un souci de proportionnalité, d’éviter d’imposer des obligations excessives en matière de cybersécurité à des intercommunalités dont la taille ne le justifierait pas. considérées comme des entités importantes les 120 communautés d’agglomération qui ne comptent pas au moins une commune de plus de 30 000 habitants, ainsi que les communautés de communes.

Morin Desailly. Cet amendement a une double visée. Premièrement, les entités concernées devront d’abord être informées et sensibilisées par les ministères concernés dans les trois ans qui suivent l’entrée en application de la loi.

Un travail d’identification croisé doit être effectué par les ministères concernés pour identifier et présensibiliser les entreprises destinataires de nouvelles obligations pour les informer et les accompagner au mieux. cet amendement vise à sécuriser les échanges d’informations et de données sensibles entre les entités concernées et l’Anssi. Il est primordial que ce partage se fasse au travers de mécanismes de protection des informations divulguées afin de garantir la confidentialité des données, potentiellement sensibles, et de les préserver d’un risque d’extraterritorialisation, conformément à l’article 31 de la loi n° 2024 449 du 21 mai 2024

M. Olivier Cadic. Les opérateurs d’importance vitale (OIV) sont désignés par les ministères coordonnateurs du secteur auxquels ils appartiennent. En cohérence, cet amendement vise à mettre l’expertise des ministères coordonnateurs des secteurs d’activité visés par l’article 7 du projet de loi au service de l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, afin que les listes d’entités importantes et essentielles prennent en compte les spécificités des écosystèmes concernés. Ainsi, certaines entités ne correspondant pas aux critères prédéfinis d’entités importantes ou essentielles pourraient être intégrées à la liste des entités concernées pour des critères stratégiques, économiques, technologiques ou sociaux relevant de l’analyse des ministères coordonnateurs. Les ministères concernés ont en effet exprimé leur souhait d’être

le texte comme un acte juridique sectoriel de l’Union, au sens de l’article 4 de la directive NIS 2, comme cela a été le cas pour le règlement Dora. Dès lors, les entités sont les plus à même de savoir si elles sont soumises

en demande donc le retrait. Quel est l’avis du Gouvernement ? Le choix a été fait de transposer l’exigence en faisant peser sur l’Anssi l’évaluation de la proportionnalité des mesures. Cette position a le mérite de ne pas rendre l’entité seule responsable de l’évaluation de son risque, ce qui pourrait la placer en difficulté,

l’avis de la commission spéciale ? La question de la sous traitance est déterminante, car le recours à un sous traitant qui serait mal protégé contre les menaces cyber peut constituer une vulnérabilité grave pour une entité. Il était donc important de faire figurer cette notion à l’article 14 du projet de loi. Je considère en revanche que les modalités précises de prise en compte de la sous traitance, notamment les rôles et responsabilités de chacun, devront être détaillées dans le décret d’application de l’article 14 du projet de loi,

La proposition de limiter la prise en compte des seuls sous traitants ayant une implication directe sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information pourrait néanmoins conduire les entités à négliger un pan de leur chaîne de sous traitance, ce qui augmenterait le risque de compromission par un acteur malveillant

de cet amendement pourrait entraîner une mauvaise transposition de la directive. En effet, si son article 21 prévoit bien la prise en compte de cette chaîne de sous traitance, elle ne restreint pas cette prise en compte aux seuls fournisseurs ayant une implication directe sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’informatique. Néanmoins, les entreprises de services numériques

les plus petites collectivités manquent souvent de ressources techniques, humaines et financières pour transposer une directive aussi importante que complexe. C’est pourquoi nous vous proposons, par cet amendement, d’étendre le délai d’application de mise en conformité à cinq ans. Ce temps permettra la mise en place de formations adaptées pour les élus, la structuration d’une filière cyber territorialisée et la mise en œuvre d’un accompagnement efficace de l’État. Accorder ce temps d’adaptation, c’est préserver l’efficacité de la directive et favoriser la montée en compétences des collectivités sur ces sujets d’avenir.

Je partage pleinement la volonté de la présidente Carrère, auteure de cet amendement, de laisser aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à leurs établissements publics administratifs

à Mme Audrey Linkenheld. Nos travaux en commission ont permis de préciser qu’un décret déterminera les conditions d’élaboration, de modification et de publication du référentiel d’exigences techniques et organisationnelles.

Cet amendement, qui tend à introduire un principe de préférence pour les entreprises de cybersécurité françaises, ne me paraît pas compatible avec les dispositions de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit la libre prestation de services.

auprès des banques, des assurances ou des clients d’une entité.

des avions de chasse, ils gardent la possibilité de désactiver à distance un certain nombre de systèmes d’armes. Il en va rigoureusement de même pour les logiciels

M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à ne pas imposer aux fournisseurs de services de chiffrement l’intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité de leur système. En effet, certaines initiatives législatives et réglementaires récentes ont cherché à imposer à ces fournisseurs l’intégration de portes dérobées (), de clés de déchiffrement maîtresses ou autres mécanismes, dont le seul but est de créer des failles exploitables par nos autorités comme techniques de surveillance. Ces sont des cadeaux faits aux acteurs malveillants – cybercriminels, États hostiles, entités privées –, comme le démontre le cas Salt Typhoon, des cybercriminels chinois ayant exploité des vulnérabilités imposées aux acteurs de la « Tech US » par le législateur américain. En outre, fragiliser la sécurité des solutions de chiffrement françaises et européennes nuirait à notre compétitivité face aux acteurs internationaux qui, eux, ne seraient pas nécessairement soumis aux mêmes contraintes. Ce projet de loi prévoit une hausse drastique des normes de cybersécurité. Où serait la cohérence si nous acceptions, dans le même texte, de créer sciemment des failles de sécurité ? Cela irait, en outre, à l’encontre des principes de sécurité reconnus à l’échelon international et imposés par la directive NIS 2.

Le chiffrement garantit une confidentialité absolue des échanges et des transactions numériques. Cet amendement a reçu un fort soutien de la part de l’écosystème cyber. Il vise à inscrire dans la loi un principe clair de sécurité numérique. Madame la ministre, comme je l’ai évoqué lors de la discussion générale,

s’agissait de renforcer la lutte contre les réseaux de narcotrafic, les groupes terroristes et, au delà, contre toutes les organisations criminelles qui tirent profit de la généralisation des messageries chiffrées et des difficultés, pour les services de renseignement, à accéder aux informations qui sont échangées

J’ai déjà eu l’occasion de rappeler mon attachement à la préservation d’un niveau élevé de chiffrement, qui est au cœur de notre confiance numérique. S’il est légitime que les autorités puissent, conformément à la doctrine nationale sur le chiffrement, obtenir, sous le contrôle d’un juge ou d’une autorité indépendante, un accès ciblé aux données,

D’une part, le chiffrement des communications, en ce qu’il concourt à la protection du secret des correspondances et de la vie privée, principe à valeur constitutionnelle, bénéficie déjà d’une première protection.

afin de permettre aux services de renseignement d’accéder au contenu intelligible des correspondances et aux données qui y transitent. Cet accès est limité aux seules correspondances et aux données ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique de mise en œuvre des techniques

enjeu de sécurité nationale. Toutes nos données, bien évidemment, sont accessibles de l’extérieur, et il est tout à fait normal que les parlementaires les protègent.

inévitablement disponibles, ou alors en chiffrant le message communiqué à l’intérieur d’une communication elle même non chiffrée. Il n’existe par ailleurs, mes chers collègues, aucune étude d’impact ni justification étayée de l’utilité de cette mesure. Un groupe de travail

en place. Bien entendu, nous voulons tous donner à nos services de renseignement la capacité de lutter contre le narcotrafic ou contre les usages criminels des messageries cryptées. Mais cela ne peut pas se

Le scrutin est clos.

Certains bureaux d’enregistrement de noms de domaine sont complices. Ils se fondent sur la confidentialité pour s’opposer à la communication des données d’enregistrement ou divulguent au titulaire du nom de domaine l’identité du demandeur de la communication de ces données. L’article 20 impose aux offices et aux bureaux d’enregistrement de conserver les données relatives à l’enregistrement des noms de domaine, sans prévoir aucune période minimale de conservation. Cette obligation demeurerait donc valable uniquement tant que le nom de domaine est utilisé. Il en résulte un risque majeur de fraude au bénéfice des délinquants numériques, qui peuvent utiliser un nom de domaine simplement durant quelques jours, avant d’en employer un autre, et en renouvelant ce processus indéfiniment, sans que l’on soit en mesure de procéder rapidement à leur identification. Pour prévenir les risques de fraude et permettre l’identification des délinquants

Cet amendement a effectivement pour objet la conservation des données relatives à l’enregistrement des noms de domaine pendant la durée d’utilisation du nom de domaine et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la cessation de son utilisation, alors que l’article 20 énonce actuellement que cette conservation n’est valable que tant que le nom de domaine est employé.

protocoles existants et de leur version modernisée et plus sécurisée, le (RADP). Ces protocoles sont standardisés à l’échelle internationale. Ils garantissent un accès simple et gratuit aux données d’enregistrement non personnelles des noms de domaine.

aux cybermenaces, laquelle renforce à son tour la capacité des entités à empêcher les menaces de se concrétiser en incidents réels et leur permet de mieux contenir les effets des incidents et de se rétablir plus efficacement. Il est donc nécessaire de permettre l’émergence, au niveau de l’Union, d’accords de partage volontaire d’informations en matière de cybersécurité. « À cette fin, les États membres devraient activement aider et encourager les entités, telles que celles fournissant des services de cybersécurité et actives dans la recherche, ainsi que les entités concernées qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, à participer à ces mécanismes d’échange d’informations en matière de cybersécurité. Ces accords devraient être établis conformément aux règles de concurrence de l’Union et au droit de l’Union en matière de protection des données. » Pour lever tout doute à ce sujet, de reprendre également le contenu du considérant 121, qui décrit le recours à la base légale de l’intérêt légitime pour fonder les traitements de données à caractère personnel qui pourraient être effectués à cette occasion et reconnaître que le partage de données concernées est conforme aux exigences du RGPD.

L’adoption de cet amendement serait donc susceptible de limiter les informations échangées entre entités régulées en matière de cybersécurité. Enfin, cette disposition viendrait ajouter des lourdeurs bureaucratiques, avec l’exigence de notification à l’Anssi

administratives et judiciaires – bref des entités de natures vraiment très diverses, allant des petites et moyennes entreprises jusqu’à différentes formes de collectivités. Il nous semble que, au regard de cette diversité, et conformément à l’esprit de l’article 21 de la directive NIS 2, il serait utile de préciser dans le texte que les mesures prescrites par l’Anssi en cas de

amendement, qui a été parfaitement présenté, vise à préciser que les mesures pouvant être prescrites par l’Anssi, lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information d’une entité, doivent être non seulement nécessaires pour éviter l’incident

du Gouvernement ? L’objectif visé par cet article est, en cas de menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes informatiques des entités visées par le texte, d’éviter la survenue d’incidents ou d’y remédier s’ils n’ont pu être empêchés. Les mesures prescrites seront donc nécessaires et proportionnées à cet objectif. L’approche de l’Anssi consiste à dimensionner ces prescriptions au cas par cas, de manière adaptée à la menace et aux nécessités opérationnelles qu’impliquent les incidents. Cela nous semble donc parfaitement cohérent avec l’amendement que vous proposez. C’est pourquoi j’émets, pour ma part, un avis favorable.

déléguée. Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 26, afin de couvrir deux situations opérationnelles. Tout d’abord, en application de la réglementation européenne et nationale sur la certification, certains certificats sont également délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité. Il apparaît donc nécessaire de prévoir la supervision de l’activité de certification desdits organismes. En outre, la recherche de manquements implique de recourir à des experts qui ne seront ni des contrôleurs au sens du premier alinéa ni des organismes indépendants. Il s’agit par exemple d’experts d’autorités de supervision d’États de l’Union européenne dans le cas d’enquêtes transfrontalières, de consultants indépendants qui pourraient faire notamment des audits, des scans, ou encore d’agents de l’État dont l’expertise pointue pourrait être temporairement utile, sans pour autant qu’il soit nécessaire de les désigner et de les assermenter

à Mme Vanina Paoli Gagin. Cet amendement tend à introduire un critère de nécessité, pour mieux apprécier et objectiver la légalité des demandes d’accès et offrir ainsi un niveau renforcé de sécurité juridique.

En tout état de cause, il est important que ceux ci puissent accéder à ces éléments, et notamment aux systèmes d’information, dans la mesure où le contrôle qu’ils mènent porte précisément sur le niveau de sécurité de ces systèmes d’information. Dans tous les cas, cet accès sera donc directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission. L’avis de

Cet amendement vise à empêcher les agents chargés du contrôle de demander à l’entité contrôlée la transcription par tout traitement approprié de ses systèmes d’information, logiciels, programmes informatiques et données stockées dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision. Je partage la préoccupation de nos collègues au sujet des capacités techniques de nos TPE et PME. Je rappelle toutefois que la complexité des systèmes d’information, logiciels et autres programmes informatiques est naturellement proportionnelle à la taille de l’entité concernée. Une telle demande, qui ne sera d’ailleurs que facultative, ne me semble donc pas de nature à constituer un obstacle insurmontable pour une petite entreprise. Je tiens également à le souligner, cet amendement tend à supprimer cette possibilité pour toutes les entreprises, y compris les plus grandes, ce qui ne me paraît pas opportun.

Cependant, nous savons tous ici que nos collectivités sont confrontées à des défis budgétaires considérables. Dans ce contexte, il serait prématuré d’ajouter des sanctions financières supplémentaires.

? Les amendements n 32 et 10 rectifié visent à permettre la communication échelonnée des informations demandées lorsqu’il n’est pas possible de les fournir en même temps. Rien ne fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées de façon progressive par l’entité contrôlée, au cours du contrôle, lorsque c’est nécessaire. En outre, je rappelle que l’amende prévue en cas de fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou de communication de pièces incomplètes ou dénaturées ne pourra être prononcée par la commission des sanctions que sur saisine de l’Anssi, laquelle disposera donc d’une marge d’appréciation.

incomplets ou inexacts ou communiqué des pièces incomplètes ou dénaturées de manière délibérée, ou bien si cette défaillance résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans le doute, le caractère répressif du dispositif risquerait donc d’être considérablement atténué, ce qui n’inciterait pas les entités contrôlées à coopérer de bonne foi aux opérations de contrôle.

Aucune circonstance ne serait en effet susceptible de justifier qu’il soit fait obstacle au contrôle de manière délibérée, notamment par la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou par la communication de pièces incomplètes ou dénaturées. Au reste, Au reste, bien que l’État dispose d’un pouvoir hiérarchique sur ses administrations et établissements publics lui permettant de leur imposer le respect de leurs obligations, il n’existe aucun dispositif similaire à l’égard des collectivités territoriales, et c’est bien normal, comme l’a souligné le Conseil d’État. Il me paraît donc justifié de prévoir la possibilité d’une amende en cas d’obstacle au contrôle, et seulement dans ce cas, la décision revenant à la commission des sanctions, laquelle disposera, comme je l’ai indiqué, d’une marge d’appréciation en la matière.

peut être le résultat d’un cas de force majeure ou de circonstances qui ne dépendent pas uniquement de la personne contrôlée. C’est pourquoi, afin de garantir une évaluation proportionnée des manquements, cet amendement vise à préciser que l’absence de coopération de la personne contrôlée doit être délibérée pour que le manquement soit caractérisé.

incomplètes ou dénaturées de manière délibérée, ou bien si cette défaillance résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans le doute, la précision proposée atténuerait le caractère répressif du dispositif et ne contribuerait pas à inciter les entités contrôlées à répondre de bonne foi aux demandes

D’autre part, elle pourrait s’apparenter à une sanction financière prononcée directement par le contrôleur, ce qui irait également à l’encontre du phasage de la procédure de sanction, tel qu’il est prévu par le projet de loi. de ces difficultés, la rédaction actuelle du texte aboutirait à une surtransposition, puisqu’elle reviendrait à faire endosser aux entités assujetties le coût des contrôles dès qu’ils révèlent un manquement, quelle que soit la nature de la mesure de contrôle utilisée pour découvrir ce dernier. Il apparaît donc que le champ d’application de cette prescription est plus large que les cas prévus par la directive NIS 2, qui ne prévoit la prise en charge par les entités du contrôle qu’en cas d’audits de sécurité ciblés.

permettrait à l’Anssi d’appliquer le principe de proportionnalité et de progressivité dans la mise en œuvre de la directive, en tenant compte, notamment, de la taille, des ressources et des efforts réalisés par l’entité contrôlée pour se mettre en conformité. Quel

Je me réjouis donc que le Gouvernement ait choisi de déposer cet amendement en séance publique. Concrètement, seul le coût des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant serait pris en charge par l’entité contrôlée, conformément aux prescriptions de la directive NIS 2, tandis que l’Anssi assumerait elle même le coût des autres types de contrôle qu’elle diligente dans le cadre de sa mission de service public. Le projet de loi initial était assez ambigu sur ce point. Or il n’est pas concevable que des entités auxquelles la loi imposera désormais le respect d’un certain nombre de normes en matière de cybersécurité doivent en plus supporter le coût des contrôles qui leur seront imposés pour s’assurer du respect des normes en question. L’avis de la commission spéciale est donc favorable sur cet amendement du Gouvernement. Les amendements n 13 rectifié et 28 visent à limiter la prise en charge par l’entité contrôlée du coût du contrôle aux cas de manquement délibéré à ses obligations. Outre qu’il est difficile, pour un contrôleur, de déterminer si l’entité contrôlée a délibérément commis un manquement ou non, il paraît préférable de modifier la rédaction de cet alinéa de façon à fixer le principe, posé par la directive NIS 2, de la prise en charge par la personne contrôlée des seuls audits de sécurité réguliers

qui décide paie ». Étant donné qu’il n’est pas permis aux parlementaires, eu égard aux règles de recevabilité financière des amendements fixées par l’article 40 de la Constitution, d’imputer les coûts induits par les contrôles à l’autorité contrôlante plutôt qu’aux entreprises contrôlées,

spéciale ? Cet amendement tend à prévoir que l’Anssi publie chaque année le montant total des coûts induits par les contrôles mis à la charge des entités contrôlées. Il s’agit évidemment d’un amendement d’appel visant à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de ne pas faire reposer sur les entités contrôlées le coût des contrôles qu’elles subissent et qui relèvent de la mission de service public confiée à l’Anssi.

Le projet de loi ne prévoit pas de date limite de mise en conformité, pas plus que de date d’entrée en vigueur des contrôles, donc des sanctions potentielles. L’Anssi a indiqué qu’elle laisserait le temps aux entités de se mettre en conformité avant d’engager les procédures de contrôle et de sanction. La mise en œuvre de la directive NIS 2 doit obéir à une certaine souplesse pour permettre aux entités nouvellement concernées d’organiser leur montée en compétences et de renforcer progressivement leurs dispositifs de sécurité, sans risquer des pénalités immédiates. Cette souplesse permettrait notamment aux entités de s’organiser,

en matière de recherche et de constatation des manquements fixe également un calendrier de mise en œuvre progressive et différenciée de ces dispositions, en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité. Comme la directive, le projet de loi ne fixe pas de date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

à ce que les premiers contrôles découlant du cadre législatif que nous sommes en train de fixer ne soient pas diligentés avant au moins trois ans de façon effective. Nous avons tenu à inscrire cet engagement dans le marbre de la loi. C’est la raison pour laquelle nous proposerons un amendement

premier alinéa de l’article 31 doit prévoir des conditions de déclenchement de la phase d’instruction compatibles avec la réalité opérationnelle des contrôles. Si c’est effectivement le cas, lorsque, de manière évidente, les mesures de contrôle ont révélé un manquement, cela doit également être possible lorsque le constat de certains faits est susceptible de révéler un manquement qui n’est pas encore qualifié ou pleinement établi au moment de l’ouverture de l’instruction. Dans certaines hypothèses, la qualification d’un manquement nécessitera des mesures d’instruction approfondies assorties de mesures de contrôle complémentaires, le cas échéant. Ainsi, la phase d’instruction permettra la qualification de certains faits au regard des réglementations mentionnées à l’article 26, justement pour déterminer si des manquements peuvent être peuvent être identifiés. C’est pourquoi il paraît important de ne pas limiter l’ouverture de la phase d’instruction uniquement aux manquements constatés et qualifiés, dans le cadre des mesures de contrôle. L’amendement Cet amendement vise à permettre l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’entité contrôlée lorsque le contrôle mené, sans aboutir à la constatation d’un manquement évident de la part de cette entité, révèle des éléments ou des faits éveillant une suspicion de manquement. Les agents chargés de l’instruction devront alors vérifier si le manquement peut ou non être qualifié et déterminer si l’adoption d’une mesure d’exécution est requise ou non dans les circonstances de l’espèce.

l’ouverture par l’Anssi d’une procédure à l’encontre de l’entité contrôlée au vu des résultats du contrôle, sans davantage de précision. De façon à encadrer l’ouverture d’une telle procédure, la commission spéciale a précisé, sur l’initiative des rapporteurs, que celle ci ne pouvait être ouverte que lorsque le contrôle révélait un manquement. Certes, dans certains cas, le contrôle n’aboutit pas à une telle constatation, mais révèle un certain nombre d’éléments ou de faits éveillant une suspicion de manquement. Il est alors nécessaire d’ouvrir une procédure pour que les agents chargés de l’instruction vérifient si le manquement peut ou non être qualifié de déterminant,

le résultat des contrôles pourra correspondre à trois états : le manquement avéré, la suspicion de manquement ou l’absence avérée de manquement. Cette troisième possibilité n’est pas qualifiable au regard des moyens mis en œuvre lors des contrôles visant à garantir plus qu’une simple conformité formelle. Dans un certain nombre de cas, des mesures complémentaires d’instruction seront nécessaires pour qualifier cette absence de manquement. Dès lors, mentionner le manquement ou la suspicion de manquement comme fait générateur de l’ouverture de l’instruction n’apporte aucune garantie nouvelle à notre sens., cela risquerait d’envoyer à tort l’idée que la réglementation présente pourrait trouver une réponse purement formelle de la part des assujettis. Il nous semble qu’il convient de conserver une procédure plus souple permettant l’engagement d’une phase d’instruction sur le fondement d’éléments plus divers : manquement avéré, suspicion de manquement, mais également besoin d’une instruction complémentaire.

de mettre en œuvre, d’autre part, doivent être adaptées à la gravité du manquement, à la taille et à la capacité opérationnelle de l’entité. Je rappelle que l’article 31 habilite l’Anssi à décider de cinq types de mesures d’exécution lorsqu’elle constate un manquement dans le cadre d’un contrôle. Elle pourra donc choisir celui qui correspond le mieux à la nature à la nature du manquement et aux caractéristiques de l’entité contrôlée. Elle pourra même clore la procédure sans adopter de mesures d’exécution lorsque la situation le justifiera. La disposition proposée ne paraît donc pas nécessaire. C’est pourquoi la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle

: La parole est à Mme Maryse Carrère. C’est le même type d’amendement que tout à l’heure. Ce projet de loi impose des obligations lourdes. Bien que la modification apportée par la commission spéciale, qui remplace l’infraction pénale par une amende administrative, soit un progrès notoire, la question de la proportionnalité des sanctions aux collectivités demeure. En effet, l’amende administrative, qui varie de 1 euro à 500 euros après deux notifications successives, permet toujours d’appliquer une majoration quotidienne en cas de retard dans la mise en conformité.

en parallèle d’une mesure d’exécution lorsque l’entité contrôlée est une collectivité territoriale, un groupement de collectivité ou un établissement public administratif appartenant à une collectivité. Bien que je partage vos alarmes sur la situation financière des collectivités, ma chère collègue, une telle différenciation entre les différentes catégories d’entités paraît d’autant moins justifiée que la mise en œuvre dans le délai imparti de la mesure d’exécution adoptée par l’Anssi s’impose à toutes les entités sans distinction. Je rappelle que l’objet d’une mesure d’exécution est non de sanctionner l’entité contrôlée, mais de mettre en terme à un manquement aux obligations qui s’imposent à elle, elle, afin d’éviter de graves conséquences pour la sécurité de ces systèmes d’information. Le fait qu’il s’agisse d’une collectivité territoriale n’y change rien. Il est donc nécessaire de prévoir une astreinte suffisamment incitative pour que ces mesures soient mises en œuvre le plus rapidement possible.

à la personne contrôlée de rendre public son manquement. Seule la commission des sanctions est désormais habilitée à décider, dans l’intérêt du public, de publier sa décision ou un extrait de celle ci. Cet amendement paraissant satisfait,

La commission des sanctions sera composée d’un membre du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes et de trois personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. Ces membres seront nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Mme la ministre déléguée. Cet amendement a pour objet la mise en conformité à la directive NIS 2 qui ne conditionne pas l’interdiction d’exercer des dirigeants des entités essentielles à la persistance d’un manquement malgré l’imposition d’amendes pécuniaires.

premier lieu, l’entité essentielle est invitée, dans un délai imparti, à pallier les insuffisances ou à satisfaire aux exigences des mesures d’exécution. En second lieu, si la mesure demandée n’est pas prise dans ce délai, l’autorité de supervision peut notamment prévoir une interdiction temporaire d’exercer pour les dirigeants, qui sont des personnes physiques, de ces entités essentielles. De plus, conformément à l’article 34 de la directive NIS 2, les amendes administratives peuvent intervenir en complément de l’interdiction d’exercer. Cet amendement vise donc à conditionner l’interdiction d’exercer des dirigeants à l’inefficacité des mesures de police administratives,

La sanction consistant à prévoir une interdiction d’exercice pour des dirigeants qui n’auraient pas rempli leurs obligations en matière de cybersécurité est très mal vécue par les représentants des entreprises entendues par la commission spéciale. Notre intention première était donc de la supprimer purement et simplement. Nous avons toutefois été sensibles au fait que, cette sanction étant prévue par la directive, sa suppression aurait présenté un risque de sous transposition manifeste. la commission spéciale, à savoir que la sanction d’interdiction d’exercice peut être prononcée en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative a été prononcée, paraît plus équilibré, quand bien même il comporterait un léger risque de sous transposition. C’est la raison

Il a déjà été question de cet amendement, qui a pour objet de prendre en compte, dans le prononcé de la sanction, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur,

le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Il va en effet de soi que toutes ces données seront appréciées. C’est pour cette raison que l’article 37 prévoit uniquement les plafonds des amendes administratives susceptibles

Il s’agira en particulier pour les 15 000 entités désormais régulées de se mettre en conformité avec le référentiel prévu à l’article 14 qu’édictera l’Anssi, ce qui nécessitera des investissements importants, le recours à des prestataires spécialisées, l’embauche de personnel qualifié, etc. Il faudra donc laisser le temps aux entités de s’organiser. C’est pourquoi il est important de prévoir des délais nécessaires avant la mise en œuvre de contrôles, de sanctions. Dans un souci de proportionnalité, ce délai est fixé à trois ans pour les entités essentielles et à quatre ans pour les entités importantes, qui sont de plus petite taille et souvent moins bien outillées pour mettre en place leurs nouvelles obligations en matière de cybersécurité. Quel est l’avis du Gouvernement ? Nous avons eu l’avis du Gouvernement ? Nous avons eu l’occasion de nous exprimer sur ce point à plusieurs reprises. Aucun délai d’entrée en vigueur autre que celui qui est relatif à la transposition par les États membres n’est prévu dans la directive. Des dispositions transitoires ou d’entrée en vigueur différée ne peuvent Ce point a été confirmé par le Conseil d’État. Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement. Pour autant, je l’ai déjà mentionné, je m’engage à ce que cette logique de progressivité soit respectée. Elle se traduira par le délai de trois ans dont j’ai parlé tout à l’heure, cours duquel les contrôles de l’Anssi ne seront que des contrôles blancs ayant une visée pédagogique et d’accompagnement. Le Gouvernement

présente le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés. Face à la menace cyber, à laquelle sont soumises maintenant quasi quotidiennement toutes les entreprises, il semble aujourd’hui pertinent de reconnaître le risque cyber comme un risque professionnel. Une cyberattaque a bien sûr des conséquences économiques pour une entreprise, mais elle a aussi des conséquences psychosociales sur l’ensemble de ses personnels. Elle crée pour ses équipes une surcharge exceptionnelle d’activité, un sentiment de sidération, parfois d’incompétence, voire de culpabilité, qui peuvent aussi entacher l’efficacité. La mise en place de nouveaux réflexes cyber après attaque peut également causer une forme de stress supplémentaire pour l’ensemble des salariés. Compléter le document unique d’évaluation des risques professionnels permettrait un engagement général de toutes les parties prenantes de l’entreprise sur cette question, puisque celles ci devraient procéder à une évaluation du risque et mettre en place une politique adaptée. Cette nouvelle obligation participerait également à l’acculturation collective au numérique du plus grand nombre, en faveur de laquelle le Sénat plaide depuis de nombreuses années. La

avons l’obligation de respecter le plus fidèlement possible la directive et de ne pas surtransposer. Nous sommes pleinement conscients des risques que vous mentionnez et de l’importance d’embarquer les employés dans la compréhension des risques cyber et la préparation à ces risques. Cependant, il nous semble qu’il s’agirait là d’une surtransposition qui ne plairait pas

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Si cette situation témoigne de l’excellence de l’expertise française dans ce domaine, il paraît indispensable de s’assurer que les acteurs privés qui bénéficient de ce savoir faire en matière de gestion de fréquences ne nuisent pas aux intérêts de la sécurité et de la défense nationale et contribuent au développement de l’économie française. C’est pourquoi les évolutions prévues à l’article 42, qui visent à accorder plus de marge à l’ANFR et au ministre chargé des communications électroniques avant, durant et après la procédure d’autorisation d’assignation de fréquences relatives à un système satellitaire, sont particulièrement bienvenues. Je pense en particulier au fait de prévoir que l’autorisation d’exploiter une fréquence ne peut être octroyée qu’à une entité de droit français ou à un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France. Le savoir faire de l’ANFR doit en effet bénéficier non à des entreprises étrangères sans lien avec la France et uniquement à la recherche de la juridiction la plus favorable à leurs intérêts, mais à des entreprises qui sont en mesure de faire valoir l’existence d’un intérêt économique ou d’un intérêt pour la défense nationale, justifiant que la déclaration soit effectuée au nom de la France. Prévoir une obligation d’établissement en France pour l’emploi ultérieur de systèmes satellitaires à des fins de fourniture de services de communication électronique poserait en revanche un problème de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit la libre prestation de services. Par conséquent, la

déléguée. Cet amendement vise à désigner la Banque de France, ainsi que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), comme autorités compétentes au titre de l’application du règlement Dora.

Adopter cet amendement serait contradictoire avec la position que nous venons de prendre sur l’article précédent.

elles doivent en priorité recourir à des prestataires qui respectent nos normes de cybersécurité, notre réglementation et notre fiscalité. Si, dans un cas précis, aucune offre n’est disponible sur le territoire, une exception peut être faite. Quel est l’avis de la commission

de vous remercier

Les plus grandes sociétés de financement exercent, pour certaines, des activités critiques pour le secteur financier français et devraient être assujetties dès la promulgation de la loi à des standards élevés en matière de résilience et de cybersécurité.

les autres sociétés de financement, de taille plus modeste, devraient bénéficier d’un report de l’entrée en application de ces exigences dans le cadre d’un calendrier de mise en conformité proportionné Cet amendement vise donc à rétablir une date d’assujettissement des petites sociétés de financement dans des délais plus adaptés, afin que, à moyen terme, l’ensemble du secteur financier français applique un niveau d’exigences cohérent.